Écologiste et Républicain entend conserver la disposition en vigueur qui prévoit que, au stade de la mise en examen, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le Fijait, résulte d'une décision expresse du juge d'instruction. Outre le fait que la mise en examen ne vaut pas condamnation, cette inscription automatique au Fijait pour les personnes mises en examen ne répond à aucune nécessité. Les personnes mises en examen au titre des infractions terroristes retenues pour le fichier soit sont placées en détention provisoire, soit font l'objet d'un contrôle judiciaire strict. Ces mesures sont, de fait, plus coercitives que celles qui résultent d'une inscription dans ce fichier. L'inscription des personnes mises en examen n'apporte dès lors aucune plus-value dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cela explique que, à ce jour, aucun juge d'instruction n'a prononcé l'inscription

garde des sceaux. Nous proposons que les mineurs de moins de 15 ans ne puissent pas figurer dans le Fijait, d'autant qu'il existe déjà un fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, lequel permet de mener des opérations de renseignement et de suivi.

un regard angélique sur l'enfance en matière de terrorisme serait une grave erreur. Trop de Français sont morts à cause de cet angélisme. Pour rappel, au Moyen-Orient, des enfants soldats âgés de 4 à 16 ans, appelés « lionceaux du califat », ont été entraînés par l'État islamique à tuer à main nue ou avec des armes. Le retour de certains de ces enfants sur notre sol ou le risque d'en voir formés chez nous constitue une menace réelle. C'est d'autant plus vrai que l'État islamique est en train de se reconstituer, avec de grands moyens humains et des infrastructures, au Mozambique. En prenant la ville de Palma cette semaine, le renouveau du djihadisme international veut créer son califat à seulement 500 kilomètres de notre frontière française de Mayotte. Notre vigilance doit être totale et notre droit adapté. En mars 2017, ce sont 56 mineurs qui étaient poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; 400 enfants et adolescents de moins de 15 ans se trouvaient en Syrie, dont 200 y seraient nés. Ce sont eux que vous voulez rapatrier, monsieur le ministre, Plusieurs dizaines d'autres mineurs sont suivis dans le cadre de mesures pénales ou civiles pour manifester des attitudes radicales, quand ils ne sont pas, de surcroît, mis en examen pour apologie du terrorisme. Plus proche de nous, ce 10 mars 2021, deux jeunes hommes de 17 et 18 ans suspectés de préparer des attentats sanglants sur notre sol, notamment contre des militaires, ont été interpellés à Mantes-la-Jolie et à Marseille. La menace islamiste est toujours présente, car aucune de ses causes profondes n'a été éradiquée. Notre vigilance ce fichier doit être renforcée, quel que soit l'âge

La générosité de nos politiques d'accueil a trop souvent été aveugle. Elle doit désormais être contrebalancée par une véritable politique d'expulsion systématique des individus dangereux. Ni complaisance ni demi-mesures, sans quoi nous ne démêlerons jamais la situation ! C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement.

que la commission a rectifiée. C'est la raison pour laquelle vous pouvez à juste titre, madame la rapporteure, parler désormais de parallélisme des formes. Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Je mets

à Mme Gisèle Jourda. L'article 3 intègre dans le fichier les infractions d'expression de terrorisme, mais sans leur appliquer les mesures de sûreté prévues pour les infractions matérielles. Nous proposons que ces mesures de sûreté s'appliquent aux personnes condamnées pour des infractions d'expression de terrorisme. En contrepartie, puisque ces infractions ne sont pas de même degré, nous prévoyons qu'elles figurent au fichier pour une durée beaucoup moins longue que ce qui est prévu pour les infractions matérielles. les personnes inscrites au titre d'une infraction d'expression de terrorisme seront retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de cinq ans pour un majeur et de trois ans pour un mineur,

est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Gold. Il est indispensable que l'usage des locaux et des salles municipales fasse l'objet d'un contrôle régulier. Nous ne pouvons courir le risque qu'ils deviennent des lieux de radicalisation en étant loués par des individus inscrits au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Ces personnes pourraient endoctriner nos citoyens avec leur idéologie répréhensible, ce qui ne peut être toléré. Il faut donc contrôler l'usage de ces lieux chaque fois que l'occasion se présente. Dans cette perspective, une solution paraît simple à adopter aux fins de limiter les risques elle consisterait à autoriser le maire à demander au préfet de vérifier si un administré le sollicitant pour la location d'une salle est inscrit à ce fameux fichier. Une fois saisi, le préfet communiquerait l'inscription ou non du sollicitant au fichier judiciaire. L'amendement n° 491, présenté

pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Le Gouvernement et les parlementaires ne veulent pas, semble-t-il, d'un pacte de sécurité partagé avec les élus locaux. Cet amendement vise à donner la possibilité aux maires d'avoir accès au fichier des auteurs d'infractions terroristes et d'y consulter les fiches des personnes résidant dans leur commune de manière habituelle ou occasionnelle, selon des modalités fixées par décret. Le maire est le premier magistrat de sa commune ; il est celui qui rend des comptes au quotidien à ses administrés et le premier à faire face à la menace terroriste. Il ne peut donc être tenu dans l'ignorance. En période de « vigilance attentat », cette mesure d'accès au fichier est une preuve de la prééminence de leur charge au service de la sécurité de leurs administrés. Trop souvent, le maire apprend dans la presse la présence d'islamistes radicalisés dans

en matière de sécurité ? Ceux qui sont en première ligne, quel que soit le combat, doivent pouvoir bénéficier de toutes les armes pour se défendre et même contre-attaquer. Aujourd'hui, les maires peuvent demander au préfet de faire un point deux fois par an sur la menace terroriste dans leur municipalité. Les élus locaux sont donc déjà dans la confidence, il convient simplement de renforcer d'autant que les menaces, tout comme les flux, évoluent de plus en plus vite dans notre monde. C'est pourquoi, mes chers collègues, les élus locaux comptent sur nous pour voter cet amendement en faveur de la sécurité locale, de la prévention des risques terroristes et de la lutte contre l'islamisme dans nos communes.

au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Ainsi, le maire pourrait mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels sa commune fait face et adapter la politique de sécurité en s'appuyant sur la police municipale et en ajustant en conséquence son déploiement et ses effectifs.

je ne suis pas fan des fichiers. Qui plus est, la généralisation de leur publication pose un véritable problème. Si ces fichiers sont divulgués aux 35 000 maires de France, qu'adviendra-t-il ? Serviront-ils,

sont destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'État dans le département, d'informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes pour certaines décisions administratives. Ces informations leur permettent de prendre des décisions de recrutement, d'affectation, d'autorisation d'agrément ou d'habilitation. Les services administratifs ou sanitaires qui sont en contact avec un public susceptible d'être vulnérable ne sont pas concernés

est l'avis du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, j'ajoute simplement à ce qu'a excellemment expliqué Mme la rapporteure que l'article 47 de la loi Informatique et libertés interdit l'utilisation d'un fichier aux fins que vous appelez de vos voeux.

Cette nouvelle infraction interroge pour deux raisons. D'une part, la notion d'« acte d'intimidation », qui est floue, ouvre des perspectives trop larges d'interprétation et ne semble pas conforme au principe de clarté et de précision de la loi pénale consacré par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

et peu accessible, puisque l'ensemble des dispositions sont déjà prévues dans notre arsenal pénal. Par ailleurs, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'interroge sur la pertinence de l'introduction d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour les étrangers. Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 4. Quel

il est prévu que toute personne qui fait pression ou exerce des menaces sur un agent de l'autorité publique ou sur un élu, pour obtenir qu'il soit dérogé, en sa faveur, à la règle commune, par l'application d'autres règles-

est particulièrement important, parce qu'il concerne la protection des enseignants. L'Assemblée nationale a fait le choix de créer, en plus du délit de menaces ou de violences instauré à l'article 4, un nouveau délit spécifique, le délit d'entrave à la fonction d'enseignant, qui vise à réprimer les pressions et insultes dont ces agents sont la cible ; c'est

cet objectif. Prenons un exemple simple. À la sortie des classes, un parent d'élève apostrophe violemment un professeur afin de lui dire tout le mal qu'il pense de sa façon de faire cours et lui intime l'ordre de modifier son discours en classe.

Cet exemple montre bien la confusion dans laquelle les magistrats risquent de se trouver, lorsqu'il s'agira de qualifier les faits. Comment distinguera-t-on les menaces et intimidations des injures et pressions ? Le risque est que, face à cette difficulté, les magistrats soient amenés à sous-qualifier les faits, c'est-à-dire à retenir le délit d'entrave, qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

que n'importe quel autre agent public, ce qui nous paraît tout à fait inconcevable. C'est pourquoi nous proposons d'intégrer le délit d'entrave de l'article 4 à l'article 4, afin que les pressions et insultes qui entravent l'exercice de la fonction d'enseignant soient sanctionnées de la même manière que tous les autres actes de menaces ou d'intimidation commis à l'encontre des agents publics. Quel est l'avis de la commission ? L'article

Bas. Monsieur le garde des sceaux, j'espère que cet amendement-ci ne suscitera aucune controverse juridique. Il s'agit simplement de prévoir que, dans le cas où une infraction est commise à l'égard d'une personne investie d'un mandat électif public, le juge peut prononcer une interdiction des droits civiques.

Boyer. L'article 4 permet au juge de prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, « soit à titre définitif, soit pour une durée minimale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue ». Cet amendement a pour objet de prévoir que le prononcé de l'interdiction du territoire français soit une obligation. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur.

On ne peut pas tout résoudre par la surenchère, me semble-t-il ; voilà ce que j'ose exprimer ce soir devant vous. La déchéance de nationalité existe,

cet amendement tend à inscrire ce principe dans la loi, à défaut d'avoir pu la faire légitimement figurer dans notre Constitution, comme le demandaient mes collègues. Cette disposition donnerait une assise juridique aux employeurs publics et privés pour lutter contre ces dérives, plutôt que de devoir s'y adapter.

indéniables, notamment l'impossibilité d'alléguer des motifs tenant à ses origines ou à ses croyances. Cela permettrait également d'éviter aux personnes de se soustraire à des contrôles administratifs ou au respect des règles de sécurité.

Cela permettrait aussi d'obtenir des adaptations particulières en matière d'application du droit du travail et, de même, cela empêcherait qu'un employeur privé ou public soit contraint de prévoir des prestations ou d'adapter des règles pour tenir compte de prescriptions religieuses auxquelles

La loi est une disposition normative qui pose une règle juridique d'application obligatoire ; elle doit donc être respectée par tous.

contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. » La commission des lois a donc

est à Mme Valérie Boyer. L'adoption de cet article à l'Assemblée nationale, à la suite, notamment, de l'assassinat barbare du professeur Samuel Paty le vendredi 16 octobre 2020, mais aussi de nombreux autres signalements, signalements, constitue une avancée nécessaire en matière de protection de nos enseignants. Ce dispositif pourrait également être étendu aux professions médicales et, plus largement, à tout agent chargé d'une mission de service public, car eux aussi peuvent être confrontés à des pressions s'ils ne se conforment pas aux

discussion commune.

cet article indique que cette liberté est conditionnée par les objectifs pédagogiques du Conseil supérieur des programmes. Or, si celui-ci a pour mission d'élaborer les programmes, c'est le ministre qui les arrête et qui diligente les instructions organisant l'enseignement. La présidente du CSP, que nous avons reçue en commission la semaine dernière, nous a bien rappelé le rôle de cette structure. La rédaction actuelle de l'article donne donc au CSP un rôle que ne lui confère pas le code de l'éducation. Aussi, il me paraît préférable de faire référence à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation, qui vise la liberté pédagogique pédagogique dans le respect des programmes, des instructions du ministre, du projet d'école ou d'établissement, du conseil et du contrôle des membres des corps d'inspection. Cette liberté est encadrée,

», répondant ainsi à une préoccupation de notre collègue députée Annie Genevard. Celle-ci déclarait en effet : « Veillons à ce qu'un professeur qui userait de façon négative de sa liberté pédagogique ne puisse pas invoquer un délit d'entrave pour justifier ce qui ne serait en réalité qu'un exercice déficient de cette liberté. »

dans le code pénal et dans le code de l'éducation, l'importance de cette liberté pédagogique qui ne peut être entravée. Le délit d'entrave

et qu'il ne cherchait pas suffisamment à traquer les séparatismes au coeur de l'école, où ils menacent la jeunesse et son éducation. De grâce, monsieur le garde des sceaux, apportez-nous une réponse un peu plus convaincante

est systématiquement au programme, elle n'est pas toujours enseignée. J'aurais souhaité que ce que nous nous apprêtons à voter s'appliquât à l'ensemble des écoles, y compris les écoles hors contrat, notamment

fait aussi partie du contrat que la Nation doit rappeler au corps enseignant et à l'éducation nationale. Nous devons garantir cette liberté, à plus forte raison quand il s'agit de transmettre des savoirs et des valeurs.

Les professeurs ne se contentent pas de lire un manuel scolaire. Pas du tout ! Ils préparent leurs cours, ils les adaptent à leur audience, qui est toujours différente.

fragilisant le corps enseignant dans son rapport aux élèves et le mettant parfois en difficulté

sont le fruit des difficultés de notre société. Dans une société qui va bien, l'école va bien ; dans une société qui va mal, l'école va mal. Depuis plus de quarante ans, le corps enseignant a parfois été laissé un peu seul sur le bord de la route. Les propositions

: La parole est à M. Fabien Gay. Cet article conforte le recours à la protection fonctionnelle pour protéger les agents publics en étendant le champ des dispositifs de signalement pour y faire entrer les atteintes volontaires à l'intégrité physique,

Il prévoit aussi que les collectivités informées d'untel risque doivent prendre sans délai des mesures d'urgence, ce qui était déjà concrètement possible et, fort heureusement, Si cet article améliore la situation actuelle en précisant les modalités de réaction aux attaques que les agents publics peuvent subir dans l'exercice de leurs fonctions, nous souhaitons raccourcir le délai permettant à un agent de savoir s'il peut bénéficier ou non des mesures de protection et d'accompagnement à la suite d'un signalement. Actuellement, l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus de la part de l'autorité compétente.

devrait selon nous être la règle. Nous proposons donc par cet amendement que l'autorité compétente soit tenue d'apporter une réponse dans un délai d'une semaine à compter de la date de signalement, et de quarante-huit heures au plus

prévoit que ce dispositif ne se substitue pas aux autres moyens d'alerte à disposition des agents, mais les complète. Dès lors, le dispositif de signalement doit s'articuler avec les autres modalités de signalements dont disposent les agents publics. La note précise qu'« il est essentiel d'organiser la circulation des informations entre les acteurs et d'articuler les réponses à donner entre les différents canaux de signalement ». C'est la raison pour laquelle nous proposons de rendre automatique l'information des représentants du personnel en cas d'activation de ce dispositif de signalement.

Concrètement, le fait pour un fonctionnaire d'avoir été victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d'intimidation devrait être pris en compte au titre des cas prioritaires de mutation, sous réserve que l'auteur des faits ait été définitivement condamné.

en l'absence de cadre législatif, de nombreuses communes, dont Lille, Strasbourg, Lyon, Nice et Toulouse, ont adopté une charte de bonne conduite que doivent signer les futurs époux et les futurs pacsés lors du dépôt de leur dossier de mariage ou de pacs. Cette charte de bonne conduite porte sur les retards de plus d'un quart d'heure à la cérémonie, le silence lors de la cérémonie, l'absence de rodéos en ville et l'absence de drapeaux étrangers dans la salle des mariages et dans les abords de l'hôtel de ville, sans que cela pose de problème particulier.

à créer un nouveau pouvoir de police permettant aux maires d'interdire les drapeaux étrangers dans les mairies et leurs abords ainsi que lors de commémorations

concilier les exigences de l'ordre public et l'exercice des libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, de réunion ou de circulation, doivent être strictement nécessaires et proportionnées

de la présence d'un drapeau qui, en soi, ne constitue jamais un trouble à l'ordre public.

Le sale boulot, c'est dire la vérité et nommer les choses. Depuis hier, nous revenons de façon récurrente sur cette nécessité de nommer les choses.

des cérémonies. Pour être tout à fait sincère, il m'est arrivé de voir quelques drapeaux arméniens, mais toujours associés au drapeau français.

Le drapeau, on le brandit comme un signe d'allégeance à la République et à la Nation. Il n'est pas acceptable que l'on se joue avec légèreté de ces symboles nationaux,

de « réglementer le fait d'arborer des drapeaux, autres que ceux de la République française ou de l'Union européenne ». Je trouve la rédaction de l'amendement tolérante. Il n'y a donc pas de raison de s'enflammer et je crois que cet amendement doit être adopté.

il est également capital d'accompagner ceux qui atteignent les 18 ans. Dans cette perspective, il nous semble essentiel de sensibiliser les jeunes devenus nouvellement majeurs tant sur la portée des valeurs républicaines, comme la laïcité, que sur l'importance de leur participation au scrutin. Aussi, cet amendement tend à instaurer une cérémonie républicaine qui se tiendra dans chaque commune, annuellement. Cet événement serait l'occasion de remettre la carte d'électeur aux jeunes citoyens et de leur présenter, avec solennité, les principes de la République à respecter. Je vous remercie

contrat d'engagement républicain, est à nos yeux un oxymore. Permettez-moi de citer Régis Debray : « Nous payons tous à présent, par une indéniable confusion mentale, la confusion intellectuelle entre l'idée de République issue de la Révolution française, et l'idée de démocratie, telle que la modèle l'histoire anglo-saxonne. En République, l'État surplombe la société. En démocratie, la société domine l'État. La première tempère l'antagonisme des intérêts et l'inégalité des conditions par la primauté de la loi ; la seconde les aménage par la voie pragmatique du contrat, de point à point, de gré à gré. » Depuis quelque temps, la loi devient une norme relative dont le sens dépend des conventions ou des contrats qui la préparent ou la mettent en oeuvre. La séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif s'estompe. Il y aurait des principes, d'une part, et des procédures de mise en oeuvre de ces principes, d'autre part. Ne seraient intangibles que les principes posés par les lois, tandis que la définition des droits issus de ces principes se résoudrait dans des procédures de négociation. Alain Supiot, professeur au Collège de France, « la du droit romain laisse alors la place à la douceur des règles conventionnelles »- la, comme on le dit en bon limousin. Avec ce contrat d'engagement républicain, madame la ministre, vous ne défendez pas la République : vous la faites reculer.

qui sollicitent une subvention publique ou en bénéficient. Sur l'initiative des rapporteurs, nous l'avons enrichi en imposant à ces structures de ne pas remettre en cause le caractère laïque de notre République. Il faut être très clair : nous refusons que les collectivités publiques financent des organismes qui contestent l'identité constitutionnelle de la France ou mènent des actions contraires à l'ordre public. Nous proposons d'ailleurs une rédaction de compromis sur ce sujet, qui pourrait tous nous satisfaire, mes chers collègues. Nous sommes ouverts à l'évolution de ce dispositif pour y inclure, par exemple, les organismes agréés par l'Agence du service civique, comme le propose fort justement Hervé Marseille. La commission a aussi très largement souscrit à l'idée de renforcer le régime de dissolution administrative des associations et des groupements de fait. Cet outil de police administrative a fait ses preuves. Nous avons cherché à mieux encadrer le nouveau pouvoir de suspension de l'activité d'une association sans aucunement nuire à son efficacité : nous y tenons.

et les objectifs visés par le texte. La commission a, pour sa part, estimé qu'il était légitime de renforcer les pouvoirs de contrôle de l'administration et que cela permettrait de ne plus allouer de financements publics à des organismes concourant au séparatisme. Même marginale, cette hypothèse doit être prise en compte. L'article 10 est ainsi en cohérence avec les dispositions de l'article 6, qui prévoit une procédure de retrait des subventions. l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, la commission a reporté d'une année l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de contrôle de régularité prévu à l'article 10 et l'obligation déclarative créée à l'article 11 pour faciliter la vie des associations. la commission a approuvé le renforcement du contrôle des financements étrangers pour les associations soumises à la loi de 1901 et les fonds de dotation. La tenue d'un état séparé des comptes permettra de mieux identifier dans leur comptabilité les avantages et les ressources en provenance de l'étranger, et de lutter contre les phénomènes d'ingérence

Cette nouvelle obligation se rapproche beaucoup d'une sorte d'autorisation préalable, très éloignée de l'esprit de la loi de 1901, qui est un texte de portée constitutionnelle, je le rappelle. L'immense majorité des associations fait vivre les principes et valeurs de la République au quotidien, au travers de leurs actions, de leur mode de fonctionnement, de leur contribution au débat démocratique et de leur rapport à la construction et à l'exercice de la citoyenneté et à la cohésion sociale. Les associations le font au plus près du terrain, au contact des réalités et de leur complexité. Au début de nos débats, j'ai évoqué le marteau qui chasse la mouche : nous y sommes ! Pour lutter contre quelques associations aux pratiques répréhensibles, le Gouvernement jette l'opprobre et la suspicion sur tout le milieu associatif. Tout cela engendrera une bureaucratie effrayante pour des associations qui ont souvent peu de moyens et peu de temps disponible. Nous connaissons tous cela dans nos petites communes. On voudrait décourager l'engagement associatif que l'on ne s'y prendrait pas autrement ... Cette lourdeur administrative n'est pourtant pas le pire aspect du dispositif de l'alinéa 5 et la notion extrêmement problématique de menace à l'ordre public à la possibilité de retrait des agréments et des subventions, c'est vers un contrôle politique des associations que l'on s'oriente. Avec cet article, ce sont toutes les actions de désobéissance civile qui seront désormais menacées, comme celles de tant de ces associations de défense de l'environnement qui oeuvrent contre les destructions commises par l'activité humaine. Demain, un gouvernement autoritariste pourrait invoquer plus largement la menace à l'ordre public pour museler, dans les grandes largeurs, l'opposition démocratique. Encore une fois, nous jouons à un jeu très dangereux, particulièrement avec cet article.

aux fondations non reconnues d'utilité publique de s'engager à respecter les principes figurant dans un contrat d'engagement républicain. Le respect de cet engagement conditionnerait la délivrance ou le maintien de la subvention publique. En premier lieu, à quoi correspond exactement ce contrat d'engagement Les dispositions contractuelles qui y figureront ne sont pas expressément énumérées. Aucune transparence ! Cela représente évidemment un problème pour nous, législateurs, alors que nous devons nous prononcer sur cette mesure. En second lieu, les associations françaises sont déjà légalement soumises aux principes d'égalité, de liberté et de fraternité. Ces nouvelles dispositions contractuelles dogmatiques et redondantes n'ont pour seul objet que d'affaiblir les petites et moyennes associations, en grande majorité vertueuses et engagées pour le bien commun, par le biais de contraintes administratives supplémentaires. Enfin, symbolique, que signifie ce contrat d'engagement républicain ? Cette mesure n'est ni plus ni moins que la matérialisation d'une logique de défiance vis-à-vis de l'ensemble des associations ; certaines, en particulier, seront désormais soumises aux interprétations arbitraires des dispositions nébuleuses de ce contrat. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoire demande la suppression de cet article. La parole

Très nombreuses sont les associations qui s'interrogent ou qui contestent ce contrat, parce qu'elles craignent une fragilisation de la liberté associative.

Que faut-il de plus ? Je considère que, dans leur immense majorité, les associations sont nos alliées pour faire respecter la République et la défendre. Pas des adversaires ! Quand on veut conduire une bataille, on soigne ses alliés et on les fédère au lieu de les stigmatiser et de les suspecter

ce contrat d'engagement républicain. Il considère en effet que les dispositions du projet de loi ne méconnaissent pas le principe de la libre administration des collectivités territoriales, dont il appartient au législateur de fixer les conditions et pour l'énoncé desquels il dispose d'une marge d'appréciation. En outre, ce dispositif n'affecte pas davantage la liberté d'association. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État ! Pour être encore plus précise, le principe de liberté d'association

relancé les emplois aidés. Mesdames, messieurs les sénateurs, si certains d'entre vous ont connaissance d'associations qui recherchent des emplois aidés et veulent s'inscrire dans ce dispositif, je suis évidemment à leur disposition pour les mettre en relation.

Les règles de la République s'imposent donc à toutes les associations en vertu de la Constitution de la République française. Point ! Nous n'avons pas besoin de contrats.

Madame la ministre, vous nous dites qu'il arrive parfois que l'on finance des associations qui mènent des actions très condamnables. Que ces associations aient signé un papier ou pas, il revient aux élus

la charte des engagements réciproques, signée en 2014 entre l'État, les représentants des collectivités territoriales et les acteurs associatifs, aurait pu ou, en tout cas, aurait dû être le cadre concret des engagements et des responsabilités. Au lieu de cela, on vient jeter la suspicion sur l'ensemble du monde associatif, voire créer un cadre juridique pour contrôler ses actions.

Elles sont les lieux où se vivent et se pratiquent les règles de la vie en société, les lieux où se fabriquent les « communs » : il existe donc d'autres chemins pour atteindre les objectifs- que nous partageons -d'une République unie autour de ses principes, des principes vivant par la volonté de tous et de toutes. Ce soir, le Sénat ne peut décemment pas

doivent vérifier, d'une manière ou d'une autre, que ces associations respectent bien les règles de droit qui ont été rappelées tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y aura une signature

mon ami Michaël Delafosse a mis en oeuvre à Montpellier un document demandant aux associations de s'engager pour les principes républicains et la laïcité.

Tout texte officiel concourant à la laïcité doit être pensé et destiné à l'ensemble des appareils religieux. La très grande majorité des croyants français se conforment aux lois de la République, mais il y a des dérives, et ces dérives il faut les contenir. Il faut traiter cela, mais il faut le faire en disant que ce n'est en aucun cas une volonté de discriminer, mais plutôt que tout le monde doit être à égalité. » À mes yeux, ce sont là des paroles sages : elles vont dans le sens de l'article 6, que, pour ma part, je voterai

Parmi les principes partagés figurent la non-discrimination des personnes, la promotion de l'égalité de la participation des femmes et des hommes dans la gouvernance et l'équilibre entre les générations et entre les milieux socioculturels dans l'exercice des responsabilités.

La République a donné naissance aux associations ; la République a donné naissance à la citoyenneté. J'ai entendu Esther Benbassa prononcer les mots « droits » et « devoirs ». La citoyenneté offre

que nous avons fait fermer, depuis 2018, 533 établissements qui s'étaient révélés être des foyers de séparatisme, qu'il s'agisse de commerces, de débits de boisson ou- je le déplore -, parfois, d'associations, dont certaines étaient subventionnées